les réserves d'usage. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie hier sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.- fin de la séance.- Débat sur la situation et le rôle de l'OTAN et sur la place de la France en son sein (demande du groupe CRCE)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre groupe a demandé ce débat sur l'OTAN au lendemain de l'offensive turque menée dans le nord-est de la Syrie avec l'aval des États-Unis. deux pays piliers de l'OTAN trahissaient ouvertement leurs alliés au sein de l'Alliance, dont la France. Cette décision américano-turque avait notamment pour conséquence le lâche abandon des Kurdes, que nous avons tous ici dénoncé.

tenu à Londres la semaine dernière et qu'a conclu une déclaration finale plus belliqueuse que jamais, adoptée à l'unanimité, ont souligné l'urgence d'un tel débat. Devant l'ampleur des défis historiques de la période, le Parlement ne peut se contenter d'être spectateur. Le Sénat s'honore de mener ouvertement cette discussion. J'espère que cela encouragera la tenue d'un débat politique de toute la société française sur des choix stratégiques pour la Nation. Les inquiétudes de notre groupe, qui étaient déjà très vives quand nous avons demandé l'organisation de ce débat, sont renforcées par les résultats du sommet de Londres. En donnant une définition de plus en plus floue et extensive de la menace terroriste, conformément aux souhaits des États-Unis et de la Turquie, en déclarant, par ailleurs, que « les actions de la Russie constituent une menace pour la sécurité euro-atlantique » et en présentant, pour la première fois, la montée en puissance de la Chine comme un défi pour l'OTAN, celle-ci, au travers de son confirme sa visée offensive, épouse les thèses de l'administration américaine et relance la course aux armements. En confirmant la mise en oeuvre de « l'initiative pour la réactivité », le secrétaire général, Jens Stoltenberg, a annoncé que, en 2020, l'OTAN serait en capacité de mobiliser, en moins de trente jours, 25 000 soldats, 300 avions de chasse et 30 navires de combat issus des différentes armées. Mais pour quelles nouvelles aventures militaires ? Là est le danger. Je dirai pourquoi, en s'enfonçant dans cette stratégie agressive, l'OTAN constitue, à nos yeux, une alliance militaire et politique unilatérale et anachronique, inadaptée aux enjeux du XXI siècle et dont il faut viser la dissolution.

En 1989, après la chute du mur de Berlin, une occasion majeure de repenser l'architecture de la sécurité collective mondiale Non seulement aucune conséquence n'a été tirée de la fin de la raison d'être historique de l'OTAN, organisation née de la guerre froide, mais la thèse de la « fin de l'histoire » a alors aveuglé beaucoup d'analystes, qui n'ont cru qu'au triomphe du système capitaliste, de son leadership américain et de son corollaire, l'extension sans fin de la domination de l'Alliance et de son bras armé. Rien n'a été perçu, à l'époque, du nouveau monde pluriel qui s'annonçait et qui est celui du XXI siècle. Aujourd'hui, dans un contexte de bouleversements inédits, de crise de l'OTAN, d'unilatéralisme américain, une seconde chance de réfléchir à ces questions se présente. Allons-nous la gâcher La lecture du monde qui nous est le plus souvent proposée, une nouvelle fois légitimée par le sommet de l'OTAN, est celle de la peur. Les attentats terroristes, éminemment condamnables et inquiétants, servent cette vision. Cette idéologie de la peur ne s'accompagnant pas d'analyses justifie une conception toujours plus belliqueuse et expansionniste de l'OTAN. Cette vision du monde est, à nos yeux, anachronique et dangereuse. Elle ignore la nouveauté des grands défis du monde actuel. Premièrement, les besoins de développement d'une partie croissante de la planète, toujours tenue en marge par le système actuel d'inégalités mondiales et par la domination de quelques pays, peu nombreux, sur la gouvernance de la mondialisation, Les soulèvements populaires survenant dans de nombreux pays montrent, d'ailleurs, le besoin d'un nouvel ordre du monde, plus juste et plus solidaire. Deuxièmement, les révolutions climatiques, démographiques et numériques appellent le partage et les biens communs, contre la confiscation des richesses par le jeu des puissances étatiques ou multinationales. Enfin, une exigence accrue de démocratie, de souveraineté et de dignité pour tous les peuples, et non plus seulement pour quelques-uns,

avant d'être une question sécuritaire et militaire, est aujourd'hui une grande question sociale. Ce n'est plus la puissance qui offre la sécurité : c'est l'inclusion sociale mondiale, or c'est elle qui fait le plus défaut. Pour avancer vers une mondialisation plus humaine, plus juste, plus respectueuse de la planète, la voie multilatérale est la seule qui vaille, contre la tentation du cavalier seul et des nationalismes

les enjeux centraux de la sécurité sont ceux de la sécurité humaine, dans toutes ses dimensions. D'ailleurs, le premier moteur des entrepreneurs de violences, terroristes, étatiques, mafieux ou prédateurs de richesses, est la misère. Nous le voyons aujourd'hui au Sahel. Comme le dit Bertrand Badie, plutôt que de relations internationales, il faudrait désormais parler de « relations intersociales » pour penser notre politique extérieure. Nous sommes au bout des logiques de puissances. Les camps, les alliances, les blocs sont derrière nous. Nous devons penser les relations internationales et de sécurité à partir d'un multilatéralisme conséquent, et non de façade, avec une ONU renforcée, avec une politique de partenariats régionaux et internationaux plus mobiles et plus fluides. L'Alliance atlantique ne nous aide pas à avancer dans cette voie ; elle nous entrave et nous confine à des politiques de confrontation toujours plus risquées. Ainsi, au moment où l'OTAN renforce son potentiel d'intervention extérieure partout sur la planète, quel bilan faisons-nous des interventions militaires menées par ses forces, en Afghanistan, au Kosovo, en Irak, en Libye, en Syrie ? Partout, des pays ravagés, la dissémination de la violence et du terrorisme, l'instabilité accrue. Où est la sécurité promise ? Au Sahel, pour les mêmes raisons, notre intervention militaire est menacée du même enlisement, des mêmes échecs, du même rejet. Quant aux politiques de développement censées prendre le relais, elles ne sont nulle part à la hauteur des défis. Le pillage économique continue. L'aide au développement piétine, alors que les dépenses militaires s'envolent.

Parlons aussi des dépenses d'armement dans le monde, dont l'OTAN est aujourd'hui le premier accélérateur, avec la politique américaine dite de « partage du fardeau ». Grâce à l'objectif des 2 % du PIB pour les dépenses militaires des pays membres, objectif insensé à l'heure où tant de besoins sociaux s'expriment, l'escalade a repris, pour le plus grand bénéfice, en particulier, des industries de défense américaines. Tous nos efforts, y compris ceux de la France, en Europe, sont tendus vers cet objectif, alimentant les dangers de prolifération- pas seulement nucléaire -que nous prétendons combattre par ailleurs. Alors que vole en éclats l'accord entre les États-Unis et la Russie sur les armes stratégiques intermédiaires, où sont les initiatives politiques de relance de la désescalade ?

Parlons enfin de nos relations avec la Russie. Le Président de la République semble décidé à engager un nouveau dialogue. C'est le bon sens, mais à quoi rime alors notre soutien sans faille à la politique d'extension sans fin du front est de l'OTAN ?

conduiront au déploiement de troupes venues des États-Unis, débarquant en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne pour se diriger vers les frontières de la Russie, en traversant l'Europe orientale. Est-ce ainsi que la France conçoit la reprise du dialogue avec la Russie ? Est-ce ainsi que la France conçoit la défense européenne ? Mes chers collègues, permettez-moi de conclure mon propos sur cette question essentielle. Le président Macron a justifié sa sortie sur la « mort cérébrale de l'OTAN » par la nécessité de réveiller les Européens. Mais pour aboutir à quoi, au juste ?

et de rendre les Américains maîtres unilatéraux des décisions stratégiques opérationnelles ? De deux choses l'une : ou la France reste embarquée dans ce projet sous leadership américain, et les lourdes questions soulevées par Emmanuel Macron resteront lettre morte, ou nous ouvrons sérieusement le débat sur un nouveau système de sécurité collective en Europe.

L'OTAN est un facteur de paix, de stabilité et de liberté pour tous ses membres, mais aussi pour les pays n'appartenant pas à l'Alliance atlantique, qui bénéficient de son effet régulateur. Il y a encore trois ans, les commentateurs comparaient l'Alliance atlantique à un point aveugle des politiques, des diplomates et des militaires français. Nous n'en sommes plus là et, si l'on peut regretter que le débat ait été hystérisé, la réflexion sur la clarification stratégique au sein de l'OTAN est, au moins, engagée. Elle était indispensable, pour trois raisons : l'évolution de la position américaine depuis une décennie au sein de l'Alliance, les dissonances stratégiques lourdes et la trop lente adaptation de l'OTAN à ces évolutions. La première cause de questionnement sur l'OTAN est le positionnement de notre grand allié, les États-Unis. Le pivot stratégique vers l'Asie, entamé bien avant l'élection de Donald Trump, se double désormais d'un désengagement américain d'une lecture commune de l'Occident. L'Europe et les États-Unis sont de moins en moins identifiés par le président américain comme incarnant un seul bloc de valeurs, réunis autour d'un même enjeu stratégique,

Nos partenaires Américains cèdent de plus en plus à une lecture purement économique de l'Alliance. Le partage du fardeau entre les États-Unis et les autres membres est légitime. Il est devenu une obsession, monopolisant les discussions lors des sommets de chefs d'État, les uns après les autres. Paradoxe ultime, alors que les Européens investissent dans leur défense, avec le Fonds européen de la défense, le secrétaire général de l'OTAN leur reproche de ne pas ouvrir les financements prévus.

Nous avons tous en tête une illustration de cette prégnance : la « clause F-35 » remplace la « clause de l'article 5 », dont la force est devenue moins évidente à mesure que le président américain laisse entendre que son application est sujette à caution. Enfin, en octobre dernier, les États-Unis, sans concertation avec leurs alliés, ont cautionné l'offensive turque dans le nord-est syrien, au détriment de nos alliés kurdes contre le terrorisme islamique. Désastre humanitaire, djihadistes étrangers libérés : cette intervention a été condamnée par la quasi-totalité des alliés. est symptomatique de divergences stratégiques de plus en plus affirmées et d'un réel enjeu de transformation de l'Alliance. La diversité des lectures des enjeux géopolitiques entre alliés ne doit plus être tue, car elle est une fragilité de l'OTAN. Nous n'avons pas, aujourd'hui, la même définition des menaces. L'Alliance, sortie de la grille de lecture de la guerre froide, peine à s'adapter aux nouvelles menaces. Qui est l'ennemi de l'OTAN aujourd'hui ? Son secrétaire général répète que, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, 80 % de la défense de l'Europe sera assurée par des pays non membres de l'Union. Mais contre quelles menaces cette défense doit-elle s'organiser ? Des divergences existent entre ceux qui ne voient la menace que sur le flanc Est

Si nous ne parvenons pas à un consensus clair en la matière, pouvons-nous accepter que, au sein d'une alliance, des marchandages tiennent lieu de politique stratégique ? Le renforcement du flanc Est a été un temps subordonné par la Turquie à l'adoption par l'OTAN de sa définition nationale du terrorisme. Ce n'est pas une attitude digne d'une alliance qui a tant à affronter. L'Alliance doit se réformer pour éviter de tels errements et garantir notre sécurité. Le commandant suprême allié Transformation (SACT), un Français, a la lourde tâche de gérer sa transformation. Notre Notre pays est ainsi l'une des forces de proposition qui tâchent de rendre plus efficaces les processus décisionnels et budgétaires du traité de l'Atlantique Nord. Nous avons là un rôle essentiel à jouer, pour que l'Alliance puisse devenir une structure plus flexible et adaptable à son environnement. Nous devons veiller à ce que ces réflexions progressent effectivement, ce qui implique une réelle appropriation du sujet par le secrétaire général, qui ne doit pas donner l'impression d'adopter systématiquement la grille de lecture du président américain. Il paraît indispensable que le Conseil de l'Atlantique Nord soit mieux informé, responsabilisé et, ainsi, à même de décider plus rapidement. La revue stratégique proposée par le Président de la République lors du sommet de Londres va dans le bon sens. Encore faut-il que nos propositions soient audibles Pour cela, chacun doit contribuer à un débat apaisé. Souffler sur les braises au lieu de souffler sur les bougies n'était sans doute pas le meilleur moyen d'endosser le rôle de facilitateur qui doit être le nôtre ! Nous ne devons pas empêcher le débat ; nous ne devons pas maintenir le. Au contraire, nous devons contribuer au récit, faire naître la discussion et partager l'effort avec nos alliés historiques, en affirmant notre puissance aux côtés et au sein de l'OTAN, pour que l'Alliance survive et perdure par conviction, et non par inertie. En conclusion, nous connaissons le prix de l'engagement pour la sécurité collective et la paix : nos soldats et les soldats du G5 Sahel morts au Mali et dans la bande sahélo-saharienne, auxquels je veux rendre hommage aujourd'hui encore, nous obligent. Nous leur sommes reconnaissants et redevables. Il importe que nous puissions partager avec nos alliés notre vision des menaces et des enjeux pour garantir la paix et la stabilité durant au moins encore

l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a bien joué son rôle de défense de l'Europe occidentale face aux appétits soviétiques jusqu'en 1989. Toutefois, depuis la dissolution du Pacte de Varsovie, en 1991, ses objectifs n'ont jamais été Les opérations conduites dans les Balkans- d'abord en Bosnie, puis au Kosovo -et celles menées en Afghanistan ont pu fournir, en apparence, de nouvelles raisons d'être à l'OTAN, et les provocations russes dans la mer Baltique ou dans l'Atlantique Nord, comme l'agression contre l'Ukraine, ont ressuscité la notion d'une menace extérieure, Poutine étant, de ce point de vue, une bénédiction pour les atlantistes qui essaient aujourd'hui de faire de la Russie une nouvelle Union soviétique, qu'il faudrait contenir. En réalité, qu'en est-il ? Certes, la Russie mène une politique agressive aux portes de l'Europe, à coups de désinformation et d'opérations obliques. Elle essaie de déstabiliser les pays européens de l'intérieur, notamment en périodes électorales, mais pas seulement. Cependant, elle reste une puissance économique dont le PIB est à peine égal à celui de l'Espagne

Certes, l'annexion de la Crimée et l'ingérence russe dans le Donbass ukrainien ont semé l'effroi dans les pays voisins. À cet égard, l'OTAN a bien fait de lancer des manoeuvres militaires dans les pays baltes. Avec leurs sanctions, les Occidentaux prennent le risque de pousser la Russie dans les bras de la Chine, mais nous ne saurions montrer la moindre faiblesse militaire face à Moscou. Pour résumer, oui, la Russie appelle la vigilance ; non, elle n'est pas une menace globale. Après Moscou, regardons vers Washington, pour prendre en la mesure d'une évolution qui ne laisse pas d'inquiéter les Européens, habitués à voir l'OTAN comme une protection irremplaçable.

Certes, le désintérêt américain pour l'Europe a plus d'une fois été démenti par l'histoire, et nous savons bien que l'investissement militaire des États-Unis sur notre continent n'a jamais été réduit et que leurs liens commerciaux, financiers et économiques

Enfin, et c'est le troisième élément de la crise actuelle de l'OTAN, un allié, la Turquie, prouve chaque jour qu'il se détache de l'Alliance par son évolution autoritaire intérieure, par son rapprochement avec la Russie- je pense notamment à l'achat de systèmes de défense russes S-400 -ou encore, récemment, par ses opérations dans le nord de la Syrie. L'attitude d'Ankara- d'Erdogan, pour être clair -a ainsi provoqué une crise politique de l'Alliance. En réalité, cette dernière n'a jamais incarné une convergence des visions du monde. Au fil de l'histoire, en dehors de la zone proprement dite du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'Europe occidentale, la solidarité politique entre membres de l'Alliance n'a jamais été évidente. Le Proche-Orient, en particulier, a toujours été un foyer de tensions majeures : je pense à la crise de Suez, en 1956, à la guerre du Kippour, en 1973, au raid contre la Libye, en 1986, et à la guerre en Irak, en 2003. La question syrienne s'inscrit ainsi dans une longue tradition et le problème de l'avenir de l'OTAN dépasse la seule question turque. La vérité est que les Européens ne peuvent pas rester indéfiniment spectateurs dans un monde instable et dangereux, où les États-Unis s'éloignent, où la Chine devient agressive, où la Russie demeure menaçante et, surtout, où la menace djihadiste ne cesse de grandir au sud de l'Europe.

En 1992, le traité de Maastricht a jeté les bases d'une politique étrangère et de sécurité commune et, en 2013, pour la première fois, un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement a été consacré à la défense. C'était une grande avancée. En 2017, une autre avancée a été enregistrée, avec la création d'une « coopération structurée permanente » par vingt-cinq États membres de l'Union européenne, pour faciliter le travail en commun.

2024. Avant d'esquisser les contours de ce qui pourrait être un jour une armée européenne, il y a une solution moins ambitieuse, mais plus réaliste : celle qui consiste à européaniser l'OTAN, pour en faire un instrument militaire capable de fonctionner en toutes circonstances, indépendamment des aléas de la politique américaine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg,

En conclusion, mes chers collègues, personne n'a intérêt à la casse brutale de l'OTAN. L'armée européenne est un beau projet d'avenir ; mais l'avenir, c'est souvent très long ... Pour faire avancer l'idée d'une défense européenne autonome, mieux vaut éviter tout raidissement de nos partenaires. Si les grands mots sont parfois nécessaires, les petits pas sont toujours plus utiles. C'est en tout cas une période cruciale qui s'ouvre pour la défense de l'Europe, une Europe qui doit savoir se décider à prendre enfin son destin en main. Face à ce nouveau grand défi qui s'offre à nous, la France se doit d'être à la hauteur du rôle historique qui a toujours été le sien dans la construction européenne. Très bien

soixante-dix ans : c'est un gage de sa solidité, certes, mais reconnaissons que la multiplication des désaccords entre partenaires, en particulier entre les plus puissants d'entre eux, la fragilise. Il faut dire que l'OTAN, pensée hier dans un monde bipolaire, à l'époque de la guerre froide, doit sans cesse s'adapter à un contexte géopolitique désormais multipolaire bien plus complexe. L'« empire du mal », comme aimait à le désigner le président Reagan, ne s'étendait auparavant qu'à l'Est. Désormais, il est bien plus diffus et se niche partout. Comme on le sait, les menaces sont multiformes : conflits asymétriques, terrorisme, cybercriminalité Soyons justes, l'Alliance sait évoluer. Elle a évolué quant à la définition de ses missions, en ajoutant à celle, initiale, de défense collective une mission de « sécurité coopérative », puis de gestion de crise, et elle mène aujourd'hui une réflexion prospective sur les questions migratoires et climatiques. Il n'en demeure pas moins que cette évolution du concept stratégique n'a de sens que si tous les États membres continuent d'avoir les mêmes attentes. Bien que la réalité géopolitique soit complexe, il importe de trouver un nouvel équilibre, devant émerger d'un dialogue constant entre ceux qui sont dans l'OTAN et ceux qui sont en dehors. S'agissant de la Russie, notre groupe a toujours prôné le maintien d'un lien russo-occidental soutenu. Cela suppose -j'ai déjà eu l'occasion de le dire -de veiller à ce que l'élargissement de l'OTAN à l'Est ne soit pas sans limite. À cet égard, rappelons que des promesses avaient été faites à Moscou au moment de la chute du mur de Berlin, et qu'elles n'ont pas été tenues ... Qu'on le veuille ou non, la Russie est un acteur incontournable pour la maîtrise des armements conventionnels ou la résolution des crises en Syrie, en Iran ou en Ukraine. Aussi le RDSE partage-t-il la position du Président de la République, qui est d'adopter une attitude plus constructive avec la Russie. La Chine est également au coeur de la nouvelle carte géopolitique en ce qu'elle constitue une grande puissance qui achète sans compter des terres en Afrique ou des ports dans le monde. Pékin ne se contente plus d'une influence régionale. Mais, là aussi, plutôt que de s'engager dans une logique de confrontation, il est souhaitable de privilégier le partenariat et la recherche d'un équilibre. La France, avec ses territoires ultramarins dans la zone indopacifique, peut être peut être une puissance d'équilibre, comme l'a exprimé le Président de la République lors de la dernière conférence des ambassadeurs. Enfin, s'agissant des pays membres de l'OTAN, j'évoquerai le cas de la Turquie, dont la capacité militaire fait un pilier de l'Alliance atlantique. On a déploré l'acquisition par ce pays de systèmes de défense antiaérienne et antimissile S-400 auprès de la Russie, tandis que sa récente intervention contre les Kurdes en Syrie nous interpelle. Si le dialogue avec Ankara doit être ferme, n'oublions pas que les Turcs ont tempéré la crise migratoire aux frontières de l'Europe en retenant 3,6 millions de réfugiés, ce qui invite aussi à des échanges ouverts. Parler de l'OTAN, c'est aussi débattre de la logique transactionnelle que pratiqueraient les États-Unis et que certains dénoncent ici parce qu'elle conduirait à la subordination de l'Europe. de l'Europe. L'abandon de souveraineté en matière de défense au profit des Américains est une réalité pour beaucoup de pays membres. La France, quant à elle, a su conserver son autonomie stratégique- c'est l'essentiel -, que garantit encore notre effort budgétaire croissant en matière de défense.

analyse. Nous devons relever plus concrètement le défi de la défense européenne. Des progrès ont été accomplis avec les nouveaux outils que sont le Fonds européen de la défense, la coopération structurée permanente ou encore l'initiative européenne d'intervention. Cependant, l'Union européenne est encore bien loin de pouvoir mener une action collective d'envergure de nature opérationnelle. Contrairement à l'OTAN, elle n'a pas encore su bâtir la matrice d'interopérabilité qui permet aux alliés d'agir ensemble. en place une capacité opérationnelle, nous devons définir nos objectifs stratégiques et rappeler quels sont les intérêts à défendre, en priorité au bénéfice de l'ensemble des pays européens, qui n'ont pas tous la même perception de la menace. À force d'être focalisés sur leur voisin russe, les pays de l'Europe de l'Est semblent considérer que l'instabilité de la zone euro-méditerranéenne est avant tout la préoccupation des seuls pays riverains de la Méditerranée. L'Europe de la défense doit incarner une puissance alternative capable de prendre ses responsabilités dans la gestion des crises qui la concernent directement, en complément de la mission de sécurité collective jusqu'alors garantie par l'OTAN. Mes chers collègues, les turbulences que traverse l'OTAN sont le reflet de celles qui agitent le monde. L'affirmation d'intérêts divergents fragilise le multilatéralisme. C'est contre cela qu'il nous faut lutter. Même si l'OTAN est imparfaite, n'oublions pas que la solidarité militaire qu'elle a mise en oeuvre nous a sans doute préservés du pire. Nul ne sait, en effet, ce qu'il serait advenu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sans cette alliance de peuples libres.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Président de la République avait souhaité que le sommet de Londres soit l'occasion d'une discussion stratégique sur le sens profond de l'Alliance atlantique,

Après avoir chassé plus de 300 000 personnes de ce territoire proche de sa frontière, l'État turc s'efforce à présent d'y installer des gouverneurs, une administration, des élus, bref

Les Kurdes sont massacrés, un véritable nettoyage ethnique est à l'oeuvre ... La Turquie incite des islamistes en provenance d'États dits « turcs » comme l'Ouzbékistan, le Turkestan oriental ou même l'Afghanistan à s'installer dans cette zone occupée de Syrie, le tout au mépris du droit international et des règles mêmes de l'OTAN. Mais nous pourrions citer les exemples de l'Afghanistan, de la Syrie, de la Libye, de l'Irak, du Kosovo, d'autres

attendant le retrait des troupes pour constituer un nouvel État islamique, encore pire que le précédent. Ne doutons pas que les atrocités, particulièrement envers les femmes, comme les exécutions publiques dans les stades, reprendraient alors. Quel est le sens de notre participation aux interventions de l'OTAN dans ces pays, sous couvert de protection des populations, si on laisse ensuite ces mêmes populations aux mains de leurs bourreaux ?

Nous en sommes aujourd'hui réduits à attendre les conclusions d'une hypothétique réunion en février entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne pour discuter des perspectives de l'Alliance.

de la seule institution où les discussions ne sont pas envisagées sous l'angle militaire. Si nous nous inscrivons dans la seule perspective de la course à l'armement, nous

la stabilité et la sécurité mondiales ne peuvent reposer sur une nouvelle institution militaire. Une Europe des peuples et de la paix : c'est cette Europe-là que nous avons voulue.

La stratégie de l'Alliance a semblé, ces derniers temps, connaître quelques flottements. Les comportements de certains membres ont pu paraître équivoques. Dès le début de son mandat, Donald Trump s'est plaint de la trop faible contribution des Européens à l'effort de défense. Il a lui-même jugé l'alliance obsolète et évoqué, en privé, la possibilité d'un retrait des États-Unis. De son côté, la Turquie a provoqué l'incompréhension de ses alliés en achetant des systèmes de défense anti-aérienne S-400 à la Russie de Poutine Poutine et en menant une offensive unilatérale contre les Kurdes de Syrie, partenaires des États-Unis et de la France contre le djihadisme au Levant. Erdogan a même indiqué que la reconnaissance, par les alliés, du caractère terroriste de la milice kurde YPG constituait un préalable à toute discussion sur les plans de défense de l'OTAN. Ces quelques dissensions ne sont pas négligeables, mais elles ne sont pas surprenantes au sein d'une organisation qui peine à réinventer sa raison d'être. L'OTAN est née à une époque où les États-Unis souhaitaient assurer la défense de l'Europe contre le péril soviétique. En soixante-dix ans, la donne a bien changé : l'Union soviétique a disparu et les États-Unis ne veulent plus assurer la défense de l'Europe. Le réveil est rude pour ceux qui ont engrangé les dividendes de la paix sans payer le prix de leur défense, car si l'Europe cesse d'être une priorité pour les États-Unis, les menaces qui pèsent sur le continent n'ont pas cessé d'exister, et de nouveaux dangers sont apparus. Il faut se rappeler que cette alliance n'a pas la même signification que l'on soit à Paris ou à Tallinn. Nous ne faisons pas tous face aux mêmes menaces et nous ne disposons pas tous des mêmes moyens. L'OTAN représente toujours, pour de nombreux États européens, la meilleure protection de leur souveraineté. À l'heure actuelle, l'Europe n'est pas en mesure d'assurer elle-même sa défense. Ce constat est forcément amer pour les Européens convaincus que nous sommes. Nous avons cependant tous le même objectif, celui de voir l'Europe protégée. L'OTAN a démontré ses capacités en assurant la sécurité de notre continent durant des décennies. Elle les démontre encore par les opérations et les exercices qu'elle conduit, souvent de façon très remarquable. Elle a permis de développer un haut niveau de coopération entre ses membres. Cependant, l'Alliance doit continuer de s'adapter aux changements des réalités géopolitiques. Le dernier sommet nous a appris qu'elle avait la volonté de traiter le djihadisme comme une menace prioritaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

La menace djihadiste n'est pas le seul changement à prendre en compte. Nos alliés Américains poursuivent leur désengagement de l'Europe et du Moyen-Orient. Les Européens n'ont donc d'autre choix que de devenir plus autonomes, comme l'a affirmé le Président de la République dans son discours de la Sorbonne, voilà maintenant plus de deux ans. Si une défense européenne forte n'a pas encore émergé, c'est bien davantage en raison de l'absence de volonté politique des États membres qu'en raison de l'existence de l'OTAN. les mentalités semblent changer. Différents projets industriels européens voient le jour et quelques États augmentent leur budget de défense. Même si les choses ne vont pas aussi vite que nous pourrions le souhaiter, elles avancent tout de même. L'OTAN peut participer à la naissance d'une défense européenne. Cette alliance nous a déjà appris que nous pouvons travailler efficacement ensemble. Tant que les membres de l'OTAN partagent les mêmes valeurs et ont les mêmes objectifs, il ne semble pas opportun de s'isoler.

Bockel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat est utile ; nous en ressentions le besoin, notamment au sein de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. j'avais d'ailleurs interpellé le Gouvernement sur les propos- excessifs et provocateurs, mais justes à bien des égards -du Président de la République, qui assurément ont secoué l'Alliance. Dans ce contexte, le sommet des soixante-dix ans de l'OTAN, qui s'est tenu à Londres la semaine dernière, a permis de mettre sur la table les divergences qui traversent l'Alliance. Deux aspects me semblent cruciaux pour l'avenir du traité de l'Atlantique Nord et pour la défense de notre pays d'abord, les questions que soulève actuellement le fonctionnement interne de la « machine OTAN », puis, plus largement, les raisons d'être de l'OTAN en 2019. Le fonctionnement interne de l'OTAN soulève trois questions. La première porte sur le partage du fardeau, mis au coeur des débats depuis la présidence Obama par les États-Unis, qui insistent sur l'importance de la participation financière de chaque État membre à notre protection collective. L'objectif annoncé et partagé est que les dépenses militaires nationales des membres de l'OTAN atteignent 2 % de leur PIB.

Cette problématique de juste contribution de chacun au financement de sa défense rejoint le débat promu par la France sur la nécessité, pour les pays européens, de travailler à notre défense commune. La dimension européenne de défense doit se renforcer, en tant que pilier européen de l'OTAN, dans le cadre de l'Alliance,

Ma deuxième interrogation est d'ordre stratégique : comment les vingt-neuf membres peuvent-ils agir de concert quand leurs intérêts politiques ou géostratégiques divergent ? Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait confiance, laquelle repose sur la clarification des priorités stratégiques de certains membres. Partageons-nous encore des valeurs et des intérêts avec M. Erdogan- et c'est un ami de la Turquie qui le dit -, qui marchande son soutien au renforcement de la protection du flanc Est contre l'adoption de sa propre définition du terrorisme Ma troisième question porte d'ailleurs sur la solidarité entre États membres, notamment quand l'un d'eux décide d'agir pour assurer la sécurité de tous. Ainsi en est-il des opérations françaises au Sahel. Contre la menace djihadiste qui prétend à la destruction de l'Occident et des valeurs que nous avons en partage, la France, avec 4 500 soldats déployés, est bien seule- hors quelques renforts logistiques bienvenus -sur un théâtre d'opérations grand comme l'Europe.

seuls. Enfin, les documents de planification de l'OTAN s'appuient sur un concept stratégique datant de 2010, qui n'a pas été récrit en 2019. La réforme des directives politiques globales n'est pas allée assez loin pour permettre d'adapter l'Alliance au XXI siècle. De ce fait, on peut aujourd'hui s'interroger surtout lorsque le Président américain remet en cause l'article 5 du traité de l'OTAN, fondement du pacte d'assistance mutuelle de l'Alliance, posant le principe de la défense collective d'un allié attaqué. Quel sens donner à l'Alliance si son principe fondateur est mis en doute par son membre le plus influent, sinon, désormais, le plus impliqué ? Le communiqué final du sommet de l'OTAN de Londres a rappelé de manière très ferme la validité de l'article 5, ce qui a permis d'affirmer, au terme d'un dialogue exigeant et franc, le souhait d'une Alliance forte et toujours actuelle. Nous le constatons tous les jours, les menaces ne portent plus uniquement sur notre continent : le champ d'action géographique, au-delà de l'Afrique, s'étend au Sud, mais aussi vers le Pacifique et le Moyen-Orient. L'Alliance doit s'interroger sur sa raison d'être : si celle-ci est de protéger l'Atlantique Nord, elle ne doit pas, pour autant, hésiter à agir aussi en dehors de sa zone de Si l'OTAN est défaillante au regard de cette nécessité absolue d'agir quand il le faut en dehors de nos frontières, alors sa raison d'être est sérieusement remise en question et son concept stratégique est sérieusement éculé. En conclusion, ce débat nous amène à nous interroger sur la triple actualité de l'OTAN et de la France électrochoc » administré par le Président de la République le mois dernier, les divergences clairement affichées par les membres de l'Alliance lors du sommet de Londres et la présence militaire française au Sahel. L'OTAN ne me paraît légitime que si elle inscrit son action

questions légitimes sur le fonctionnement de l'Alliance et sur ses raisons d'être que se posent ses membres ne doivent pas nous paralyser : elles doivent au contraire être une force motrice pour redynamiser notre traité, pour lui redonner tout son sens dans un monde qui n'est plus celui de la guerre froide. Cela ne sera possible que si les États membres discutent entre eux, réaffirment leur position, notamment envers la Turquie, car les alliances ont toujours autant à craindre de l'intérieur que de l'extérieur. C'est à ce prix que nous éviterons la dislocation de la plus grande alliance militaire de défense commune que le monde ait jamais connue et que nous pourrons espérer prolonger la plus longue période de paix que l'Europe ait vécue,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au côté de la chapelle du cimetière de Colleville-sur-mer, où reposent 10 000 jeunes Américains tombés pour libérer la France et l'Europe de la barbarie, on peut lire l'inscription suivante : « Leurs tombes sont le symbole éternel de leur héroïsme et de leur sacrifice à la cause commune de l'humanité. La relation transatlantique, qui est à la genèse de l'OTAN, est ancienne. La fraternité d'armes entre la France et les États-Unis remonte à leur indépendance, au XVIIIsiècle, fraternité jamais démentie et ô combien renouvelée au cours de la Première et de de la Seconde Guerres mondiales. Mais, comme le rappelle de façon touchante et juste l'inscription que j'évoquais, notre combat commun est plus qu'un engagement militaire : c'est un combat pour des valeurs communes. La primauté du droit sur la force ; la défense de la liberté des individus et des peuples ; le respect de la personne humaine : l'OTAN a été construite sur ces valeurs, au-delà de la solidarité totale entre les alliés si l'un d'entre eux était attaqué. Bref, l'OTAN est autant un outil militaire qu'un concept politique, celui d'une communauté de pays ayant des visions du monde convergentes. La France n'a pas dit autre chose lors du sommet de Londres. Certes, l'intervention du Président de la République a été particulièrement vive, mais elle était nécessaire. Ces derniers temps, temps, l'OTAN paraissait s'être réduite à une structure logistique et comptable, où l'apport de chacun n'était mesuré qu'en termes de dépenses d'équipement, en particulier si ces dépenses permettaient d'acheter du matériel au principal contributeur, dans un partenariat qui semblait devenir toujours plus commercial. Depuis l'effondrement du rideau de fer, l'horizon politique et géostratégique de l'OTAN s'est brouillé. Pourtant, c'est sur l'Alliance atlantique que la sécurité de l'Europe repose aujourd'hui. Mais pour qu'elle garde tout son sens, il faut qu'elle intègre les menaces d'aujourd'hui. La première question, qui, en réalité, n'est plus pensée depuis la chute du mur de Berlin, est celle de l'architecture globale de sécurité en Europe. Pour la traiter, il faudra parler avec la Russie, avec bien sûr la fermeté nécessaire et sans naïveté, mais sans dogmatisme, comme nous le faisons au Sénat. Les Européens doivent être parties prenantes à cette architecture, qui peut d'autant moins se limiter à un dialogue entre les États-Unis et la Russie que les États-Unis n'entendent plus assumer la même part dans la défense de notre continent. C'est pourquoi il faudra que le rôle des Européens dans leur propre défense soit au coeur des travaux du groupe de réflexion mis en place au sein de l'OTAN après le sommet de Londres. L'Alliance atlantique sera forte si elle repose sur deux piliers forts, un de chaque côté de l'Atlantique. C'est ce que nous devons faire pleinement accepter à nos amis Américains. C'est aussi ce que nous devons faire comprendre, parfois, à nos amis Européens. deuxième axe de réforme de l'OTAN tient à l'analyse des menaces. Aujourd'hui, les pays européens sont menacés par le terrorisme ; la France vient une nouvelle fois de payer le prix du sang. Pour que l'Alliance soit en mesure de répondre à ce défi, il faut une analyse partagée de la menace. Il est clair que nous n'avons pas la même définition du terrorisme que nos alliés Turcs, Le positionnement de la Turquie devra donc être clarifié sur cette question, mais aussi sur les relations avec les autres alliés, en particulier la Grèce ou Chypre. Il faudra aussi examiner, cela a été dit, les conséquences de l'acquisition de systèmes de missiles S-400 russes par la Turquie, qui soulève tout de même un problème conceptuel. Sur tous ces sujets, il est indispensable que les pays européens avancent ensemble. Nombre de nos partenaires connaissent des évolutions rapides de leur scène politique : on vote aujourd'hui même au Royaume-Uni ; en Allemagne, l'équilibre de la coalition semble incertain ; en Italie, une nouvelle coalition est au pouvoir À nous, Européens, de nous adapter à ces changements et de trouver les voies- sans arrogance, du côté français ! -pour avancer ensemble, pas à pas, pour construire, « brique après brique », une véritable défense européenne. Il faudra enfin prêter une écoute et une attention particulières à nos alliés Baltes, d'Europe centrale et orientale, souvent inquiets de notre volonté de rouvrir le dialogue avec la Russie. Ce travail de refondation de l'OTAN et de réveil stratégique européen peut être salutaire s'il est une étape dans la construction d'une défense européenne renouvelée, reposant sur un pilier transatlantique et sur un pilier proprement européen, reflet de l'autonomie stratégique européenne. Mes chers collègues, jamais le monde n'a été aussi dangereux, jamais il n'a été aussi instable. La première garantie que nos concitoyens attendent de l'État, c'est la sécurité. Soyez persuadé, monsieur le ministre, que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat sera à vos côtés pour travailler en ce sens. Faisons en sorte d'imaginer ensemble cette nouvelle architecture de sécurité de l'Europe,

Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, une semaine après le sommet de Londres, je suis très heureux que le Sénat ait souhaité se saisir de la question du devenir de l'OTAN.

et au débat stratégique et politique qui s'est engagé sur cette base avec nos alliés de l'Alliance atlantique. Nous sommes partis d'un constat, auquel nombre des interrogations que vous venez de soulever, les uns et les autres, font écho l'Alliance se trouve dans une situation de trouble politique. Les manifestations de ce trouble sont claires. Il y a d'abord un enjeu de confiance sur la force de la relation transatlantique.

un retrait du nord-est syrien, à la suite de l'offensive engagée par la Turquie, a créé un trouble. L'ensemble de ces éléments constitue un changement de nature stratégique, dont il faut tirer les conséquences.

y a, enfin, un enjeu de responsabilité, car nous observons, outre les facteurs que je viens d'évoquer, que l'environnement stratégique dans lequel évoluent les Européens est rendu plus complexe

de défense ou d'opérations, pour assumer davantage de responsabilités dans le contexte transatlantique que j'ai décrit. C'est pour toutes ces raisons,

Elle s'est incarnée dans des discussions que le Président de la République a eues d'abord avec le président Trump, puis avec le président Erdogan, conjointement avec la Chancelière allemande et le Premier ministre britannique. Elle s'est bien évidemment poursuivie dans le cadre de la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, qui a rassemblé les chefs d'État et de gouvernement, le 4 décembre.

Le premier enjeu, c'est la définition des finalités stratégiques de l'Alliance, qui implique, plusieurs d'entre vous l'ont dit, d'avoir une vision partagée des risques et des menaces. En d'autres termes, qui est l'ennemi ?

il nous faut aboutir à une analyse partagée de la définition des finalités stratégiques. Le Président de la République l'a rappelé lors de sa conférence de presse finale à Londres, la Russie la Russie constitue une menace : c'est une réalité que nous constatons dans le domaine cyber, et elle peut l'être aussi dans dans son voisinage, comme la crise ukrainienne l'a montré. C'est bien la raison pour laquelle l'Alliance a mis en place une posture de dissuasion et de défense renforcée, à laquelle la France participe pleinement. Mais la Russie est aussi un voisin sur le plan géographique et un partenaire potentiel. Nous devons donc la traiter comme telle, en assumant un dialogue de confiance et de sécurité avec elle, sans naïveté ni complaisance. C'est le sens de l'initiative en faveur de d'un climat de confiance prise par le Président de la République lors du sommet de Brégançon avec le président Poutine. Nous savons par ailleurs que la montée en puissance militaire et technologique de la Chine impose une réflexion stratégique. Toutefois, ce pays n'est pas l'objet désigné de notre défense collective

au Levant comme au Sahel. Pour cela, il est urgent que nos alliés s'impliquent davantage. Cela ne signifie pas automatiquement que l'OTAN en tant qu'organisation doive prendre des initiatives, mais les alliés qui la composent savent bien

; enfin, chacun des pays concernés doit prendre les engagements politiques nécessaires, en particulier pour la mise en place de l'accord de paix au Mali.

Ce que nous appelons, en Europe, l'autonomie stratégique, que nous devons renforcer, recouvre en fait une conception élargie du partage du fardeau invoqué par notre allié américain. C'est aussi un partage de la responsabilité. C'est le sens des initiatives que nous prenons dans le cadre de l'Europe de la défense.

La contribution de l'Union européenne doit prendre plusieurs formes. Les Européens doivent se saisir des grands sujets stratégiques concernant directement leur sécurité, dont la reconstruction d'un agenda et la mise en oeuvre de mesures tendant à la maîtrise des armements. Il faut, sur ce sujet, reconstruire un cadre de droit et appliquer des mesures de transparence pour limiter les risques d'escalade involontaire et fixer des contraintes sur les capacités de nos adversaires potentiels.

que l'Europe puisse intégrer cette nouvelle donne et fasse de cet anniversaire le moment d'une relance de l'architecture européenne de sécurité collective.

davantage de consultations de nature politique. Les discussions avec la Turquie qui ont pu se tenir à Londres ont évidemment porté sur cette nécessaire coordination. Un allié ne peut pas intervenir militairement contre nos partenaires dans le combat contre Daech, alors même que nous luttons conjointement contre les groupes terroristes.

le Président de la République a marqué sur ce point sa solidarité à l'égard de notre allié grec, à la suite de la signature de l'accord entre le gouvernement libyen et la Turquie, qui suscite des préoccupations fortes et légitimes. est l'agenda de la réflexion stratégique que nous nous sommes donné et sur lequel les chefs d'État et de gouvernement ont pu échanger lors du sommet de Londres. À l'issue de ce sommet, je constate que nous avons obtenu des résultats significatifs. D'abord, je le répète, la réflexion stratégique est engagée.

proposé par les ministres des affaires étrangères au printemps de 2020, puis à des propositions concrètes. Ensuite, nous avons rappelé clairement la solidarité de la France à l'égard de nos alliés de l'OTAN.

Ce dialogue doit permettre de défendre les intérêts de tous les Européens, sans négliger les intérêts de sécurité de nos partenaires, car ce sont aussi les nôtres. Ce dialogue doit permettre d'avancer sur un dossier comme celui de l'Ukraine. Nous l'avons vu lundi dernier, avec la tenue à Paris d'un nouveau sommet au

S'agissant de notre relation avec la Turquie, les discussions que nous avons eues ont permis des clarifications. Sur la question du terrorisme, nous n'accepterons pas que notre partenaire, le PYD, avec qui nous continuons le combat contre Daech dans le nord-est syrien, soit qualifié d'organisation terroriste.

de la Russie avec les capacités des autres alliés de l'OTAN. Cette compatibilité est bien évidemment un atout et l'une des forces de l'Alliance. Enfin, je crois que notre message sur la nécessité, pour les Européens, d'être plus responsables et plus capables au sein d'une alliance refondée et rééquilibrée, a pu être exprimé avec force et sans aucune ambiguïté. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la contribution que je voulais apporter au débat dont vous avez pris l'initiative. Nous sommes au début de cette réorientation stratégique, et nous aurons l'occasion, au cours des semaines à venir, de

en son sein. Je n'ai été saisi d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents. Elles sont donc adoptées.